L’ordre du jour appelle la désignation des vingt trois membres de la commission d’enquête sur les politiques publiques face aux opérations d’influences étrangères visant notre vie démocratique, notre économie et les intérêts de la France sur le territoire national et à l’étranger, afin de doter notre législation et nos pratiques de moyens d’entraves efficients pour contrecarrer les actions hostiles à notre souveraineté ; et des dix neuf membres de la commission d’enquête sur la paupérisation des copropriétés En application de l’article 8 , alinéa 5 de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions orales. La parole est à M. Pierre Jean Verzelen,

Cette trajectoire de hausse a été programmée, à ce stade, jusqu’en 2025. Elle est associée à des contreparties financières, pour les collectivités comme pour les entreprises qui engagent des projets industriels de tri et de recyclage des déchets, de manière à les accompagner dans l’évolution des pratiques.

renforcement, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, des coûts pour les metteurs sur le marché, de manière, là aussi, à fluidifier, mais aussi à moraliser le dispositif. le renforcement des soutiens financiers versés aux collectivités pour les tris des emballages ménagers a conduit à les faire passer de 750 millions d’euros en 2022 à 1,2 milliard d’euros en 2024, soit

retenait alors comme base de calcul le produit attendu connu, soit environ 11 milliards d’euros. Plusieurs modalités de reversement ont été mises sur pied. En apparence, la promesse d’une compensation de la CVAE à l’euro près semble respectée. Mais qu’en est il en pratique ?

les modalités de reversement retenues, notamment le recours au fonds vert, pensé alors comme un mécanisme de compensation fondé sur une dotation. Toutefois, sa répartition étant pilotée par le préfet de département au gré des projets déposés par les communes, le fonds vert ne garantit aucunement une dotation individuelle à chaque commune. Il ne constitue donc pas une ressource propre au sens de l’article 72 2 de la Constitution. Ainsi, nombre de communes et d’intercommunalités, notamment rurales, n’ont pas touché un seul centime issu de ce fonds et n’ont donc pu bénéficier d’une compensation à l’euro près.

la CVAE ne varie pas de manière homogène partout sur le territoire, puisque, à la différence d’un certain nombre de paniers de fiscalité, elle repose sur le dynamisme réel des bases locales, et elle est locales, et elle est totalement cyclique. Elle peut baisser, à la différence de la taxe professionnelle – cela a fait partie des raisons pour lesquelles le mécanisme que je vous ai présenté a été retenu. Il peut donc y avoir, au sein d’une progression nationale, des baisses localisées.

des territoires. Monsieur le ministre, le transfert de la gestion des digues domaniales par l’État est prévu par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi Maptam.

En atteste la collaboration entre l’Établissement public Loire (EPL) et la création d’une plateforme à Tours. Cependant, des difficultés majeures émergent, notamment concernant la convention de fin de gestion entre l’État, l’EPL et les établissements publics de coopération

En outre, la contrainte imposée aux EPCI de délibérer sur cette convention avant le 28 janvier 2024 sans disposer d’une version stabilisée du projet soulève des inquiétudes légitimes. Cette situation place ces établissements publics face à un dilemme : présenter une version non aboutie ou organiser un conseil extraordinaire, avec un risque politique qui est, comme chacun le sait, La charge financière imposée aux EPCI, sans compensation adéquate de la part de l’État, est particulièrement préoccupante. Cette charge affecte directement le budget des actions locales essentielles. En cette période de crise,

ferrée à grande vitesse – j’y reviendrai. Cette décision est brutale, car elle n’a fait l’objet d’aucune concertation ni d’aucune information, alors même que l’offre est aujourd’hui réduite et après que les contribuables, dont les Azuréens, ont servi d’assurance vie face aux crises covid. Enfin, cette décision est lourde de conséquences. Vous le savez, monsieur le ministre, je défends le ferroviaire, mais je pense qu’il faut le bon mode de transport au bon endroit. Aussi, qu’entendez vous faire pour que la compagnie nationale Air France revienne sur sa décision ou renonce à toute dégradation de l’offre

Le trafic de la navette Orly Nice a diminué de 60 % par rapport à 2019. La clientèle affaires est passée de 100 000 passagers en 2019 à 50 000 en 2023.

Cela dit, je vous rejoins sur un certain nombre de points, en particulier sur le fait que ces évolutions ne doivent pas se faire au détriment des territoires et de leur connectivité. En outre, vous avez raison, le nombre de rotations, la manière dont les choses se passeront et la façon dont Air France continuera à assurer un service constituent

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous savons combien la rénovation énergétique est une priorité pour nos objectifs climatiques, pour les enjeux

des citoyennes, des citoyens et des élus locaux se sont constitués en collectif d’associations, pour interpeller les décideurs et alerter sur les risques qui accompagnent le projet Depuis plusieurs années, ils se mobilisent pour porter un projet de substitution. Ils ont déposé plusieurs recours, soutenus par les élus locaux, y compris par ceux de la majorité présidentielle, et par de nombreux agriculteurs, très inquiets pour leur production et la pollution de leurs terres.

Ensuite, vous faites état d’une contestation locale, ce qui correspond à une réalité, mais la validation de ce projet, à l’issue d’une procédure longue et pour laquelle je ne suis d’ailleurs pas totalement certain que l’intégralité des recours et des procédures ait d’ores et déjà été évoquée,

qui a été mis en place. D’après le Gouvernement, 22 000 communes devaient être concernées par ce filet de sécurité inflation, une aide qui était, vous le savez, monsieur le ministre, particulièrement attendue par les élus locaux dans un contexte de hausse du coût de l’énergie dont les conséquences sont lourdes

Le Gouvernement a appliqué les critères qui ont été votés par le Parlement. Si vous regrettez que nous ayons respecté ce qui a été voté par la représentation nationale, nous devons tous reconsidérer notre rôle et notre place dans cet hémicycle

ont reçu une aide alors même qu’elles n’en avaient pas le droit. Cela a été le cas de 2 527 communes, pour un montant de 68 millions d’euros – à rapprocher des sommes que vous avez évoquées plus tôt. Dans l’absolu, c’est une bonne nouvelle : cela veut dire que la situation a été moins grave que ce qui avait été anticipé, et par le Gouvernement, et par le Parlement. Les reprises d’acomptes portent très majoritairement – dans 75 % des cas – sur des montants inférieurs à 10 000 euros. Elles sont

sur les 40 communes que compte mon département, 38 sont classées en zones d’intervention prioritaire par l’agence régionale de santé (ARS). En Seine Saint Denis, de nombreux habitants ont été en première ligne lors de l’épidémie de covid 19. Ils ont été honorés pour leur présence sur le terrain.

J’attire votre attention sur cette situation, monsieur le ministre, parce qu’elle constitue bien plus qu’une double peine au regard de la défaillance du droit commun sur ce territoire. Je tiens à rappeler que, loin des préjugés qui ont la vie dure, la Seine Saint Denis n’est ni un puits sans fond pour l’État, ni un territoire gâté de la République. La réalité, c’est qu’il s’agit du troisième département contributeur national à la TVA et du huitième pour ce qui concerne les cotisations sociales. Pourtant, en retour, la politique de la ville ne parvient pas à pallier le déficit de droit commun ; en retour, la Seine Saint Denis constitue le premier désert médical de France.

la capacité de l’État à proposer à de nouveaux médecins de s’établir prioritairement dans les zones en tension : comment faire pour que ces médecins puissent s’installer dans les quartiers prioritaires, ce qui constituerait une mesure d’équité pour l’accès à la santé ? La parole est à M. le ministre. Monsieur le sénateur

Dans la continuité du plan de transformation des Ésat, la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi apporte des avancées concrètes pour rapprocher les droits des travailleurs en situation de handicap de ceux des salariés le remboursement des frais liés aux transports publics, l’accès aux titres restaurants et aux chèques vacances, la prise en charge à 50 % de la couverture complémentaire collective vont améliorer la situation de ces travailleurs, de même que l’augmentation de la rémunération directe, à hauteur de 15 % du Smic, qui est envisagée. si ces nouveaux droits contribuent légitimement à l’amélioration de leur statut, ils représentent aussi des coûts supplémentaires pour les Ésat, alors que la situation financière de ces derniers est déjà particulièrement complexe. Aux termes d’une enquête flash d’octobre 2023 menée par le réseau Unapei, en lien avec d’autres organisations, et à laquelle près de 500 structures ont répondu, 27,5 % des Ésat du réseau Unapei sont en déficit net. Par ailleurs, selon l’Observatoire économique national des achats responsables, 31 % d’entre eux sont à l’équilibre ou excédentaires de moins de 50 000 euros. Avec le financement de ces nouveaux droits, la majorité des Ésat risque de se trouver en situation de déficit, alors que ce modèle est le seul qui permette l’emploi des personnes avec d’importants besoins d’accompagnement. Le soutien de l’État est donc indispensable. Je le rappelle, les Ésat sont des lieux d’accès au travail essentiels pour plus de 120 000 personnes en situation de handicap, qui y sont encadrées et accompagnées spécifiquement. Aussi, partageant les inquiétudes relatives au devenir de ce modèle, je souhaite connaître les actions que le Gouvernement compte prendre pour compenser ces nouvelles dépenses et afficher son soutien. La parole est à M. le ministre.

au lieu d’être placés dans une situation spécifique. La loi pour le plein emploi de novembre 2023 a d’ores et déjà élargi à ces travailleurs l’accès à la couverture complémentaire santé et au remboursement des frais de transport, ainsi que l’accès aux chèques vacances et aux titres restaurants.

les tribunes. L’ordre du jour appelle l’examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales. Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix.